Mme Angèle Préville. Lors du scrutin n° 101 sur l'amendement n° 120 rectifié tendant à rétablir l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République, ma collègue Gisèle Jourda a été enregistrée comme votant pour, alors qu'elle ne

: La parole est à M. Pierre-Antoine Levi. « Une école qui ferme, c'est un village qui meurt. » Dans les communes rurales, la décision de fermer une école a des conséquences dramatiques pour les habitants de la commune, mais aussi pour les élus. La loi contraint les communes à financer le fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association avec l'État, notamment les dépenses de fonctionnement relatives au transport des élèves lors des activités scolaires, à la médecine scolaire, à la rémunération d'intervenants lors des séances d'activités physiques et sportives et aux classes de découverte.

Cet amendement vise les financements d'organisations ou d'États étrangers, car ils peuvent donner lieu à une ingérence de puissances étrangères dans les activités éducatives françaises. Il convient donc de restreindre la communication des informations budgétaires et comptables à ces seuls financements.

monsieur le ministre,

la protection de l'enfance et de la jeunesse, mais aussi que les enfants soient dans un environnement leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires au socle commun. Néanmoins, le fait que ces établissements soient prévenus en amont de ces contrôles- j'ai déjà

Quel est l'avis de la commission

La parole est à M. Max Brisson. Cet amendement vise à ce que les résultats des contrôles diligentés dans les établissements hors contrat exposent précisément les explications et les améliorations que le directeur doit

explicitement que « la mise en demeure adressée au directeur de l'établissement doit exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l'enseignement dispensé soit mis en conformité avec l'objet

l'avis du Gouvernement ? Les résultats du contrôle sont notifiés à l'établissement dans les conditions fixées par l'article L. 442-2 du code de l'éducation, avec l'indication du délai dans lequel il est mis en demeure de fournir ses explications et d'améliorer la situation. L'exigence de motivation a d'ores et déjà été rappelée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 1 juin 2018. Il est ainsi précisé que les mesures nécessaires pour que l'enseignement dispensé soit mis en conformité avec l'objet de l'enseignement obligatoire doivent être exposées à l'établissement de manière précise et circonstanciée. Les académies ont reçu pour instruction de se conformer à cette réserve constitutionnelle par le biais d'une circulaire du 21 août 2018. Dans le cadre des formations délivrées par les services centraux du ministère, cette exigence est toujours rappelée. L'amendement étant satisfait, j'en demande le retrait.

d'un strict point de vue juridique. Nous savons que l'école Al-Badr de Toulouse, qui a fait l'objet de plusieurs décisions de justice, dont une de fermeture, a vu cette dernière annulée parce que la décision était insuffisamment motivée.

fixant à un mois le délai au cours duquel le directeur de l'établissement doit régulariser sa situation à la suite d'un contrôle. Il permet ainsi de prévoir un délai suffisant, prévisible et identique d'une académie à l'autre. Toutefois, afin de prévoir les situations d'urgence, c'est-à-dire dans les cas de « risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement » et de « manquements aux obligations en matière de contrôle de l'obligation scolaire et d'assiduité des élèves », cet amendement prévoit qu'un délai plus court pourra être fixé par l'administration pour agir rapidement. Cette mesure doit permettre à l'administration d'utiliser

M. Max Brisson. Les contrôles diligentés par l'éducation nationale ne doivent pas concourir à aligner les progressions, les programmes, les supports et les méthodes scolaires des établissements privés hors contrat sur la pratique de l'éducation nationale. Les contrôles doivent bien porter sur les insuffisances de l'enseignement par rapport aux objectifs de l'instruction obligatoire et à l'acquisition progressive du socle commun de connaissances et de compétences, et non sur la manière dont les programmes sont traités, les progressions définies et les méthodes fixées. ... Quel est l'avis de la commission Même si ce socle commun est bien transmis, certains contrôles remettent en cause les choix pédagogiques des établissements. Cet amendement de Max Brisson vise à garantir la liberté pédagogique des établissements privés hors contrat. À ce titre, la commission y est favorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? La question La question soulevée par cet amendement trouve déjà une réponse dans les textes en vigueur, qui assurent le respect de la liberté et de la spécificité pédagogiques des établissements privés hors contrat. de l'article L. 442-3 du code de l'éducation, les établissements scolaires hors contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques. Par ailleurs, l'article R. 131-12 du code de l'éducation prévoit que, dans les établissements hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences doit être progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le respect de ces éléments est d'ailleurs régulièrement rappelé aux équipes d'inspecteurs lors des sessions de formation sur les établissements hors contrat qui leur sont proposées. Le Gouvernement estime que l'amendement est satisfait.

à l'inspecteur d'académie, représentant de l'État dans le domaine de l'éducation nationale, d'exercer un contrôle sur les établissements privés qui ne sont pas liés à l'État.

universelle, c'est-à-dire pour l'ensemble des établissements de France, l'égalité entre les femmes et les hommes et les enjeux de la mixité- nous sommes bien d'accord sur ce point. Le droit actuel

Vous avez parfaitement compris le sens de mon amendement, monsieur le rapporteur pour avis. Relisez-le : je ne demande pas l'interdiction de l'enseignement non mixte,

Je suis désolé de vous le dire, mais, dans certains établissements, il y a une fabrication sociale du genre. On transforme des petites filles en femmes, et des petits garçons en hommes par

dans les compétences très larges de l'inspecteur d'académie une mission particulière sur la mixité. Avec le temps que nous avons consacré à la libération des femmes la semaine dernière, je ne comprendrais pas, mes chers collègues, que vous ne puissiez pas voter cet amendement, puisque vous partagez notre souci universaliste de l'émancipation féminine.

du code de l'éducation déterminent les cas d'incapacité d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement au sein, respectivement, d'un organisme privé d'enseignement à distance, d'un organisme de soutien scolaire

Cette incapacité se traduit par l'obligation, pour l'employeur, de s'opposer à un recrutement ou à une nomination ou, s'il s'agit d'un agent en exercice, de mettre fin à ses fonctions.

911-5 du code de l'éducation. Dans un souci de cohérence et afin de lever toute ambiguïté, le présent amendement a pour objet d'étendre la précision apportée par l'article 22 du projet de loi aux articles L. 444-6, L. 445-1 et L. 731-7 du code de l'éducation. Quel

doit exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l'enseignement dispensé soit mis en conformité avec l'objet de l'instruction obligatoire ». Du reste, le Sénat a inscrit ce principe dans la loi,

Enfin, le code pénal punit actuellement d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas prendre les dispositions nécessaires pour que l'enseignement dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire.

concerne les établissements privés hors contrat déjà installés, les inspecteurs académiques spécialisés du département dont je suis élue m'ont confié qu'une injonction de fermeture pouvait prendre jusqu'à trois ans. Le régime de fermeture administrative proposé dans ce texte est donc très attendu sur le terrain et le renforcement des sanctions à l'encontre des chefs d'établissement d'enseignement privé hors contrat ignorant les différentes mises en demeure ou la demande de fermeture est, dans l'idée, bienvenu. le montant des amendes n'aura, je pense, que peu d'impact face à des insolvabilités souvent organisées. C'est pourquoi cet amendement vise à ce que le juge interdise aux directeurs d'enseigner ou de diriger un autre établissement scolaire, en cas de non-respect des obligations prévues par la loi. Cela nous permettrait d'économiser beaucoup d'énergie ; fermer une école pour qu'en ouvre une autre, avec la même direction, quelques mètres plus loin, n'a aucun sens ...

Le juge pénal en fixe la durée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce. Dans la pratique, les peines complémentaires n'ont été prononcées par le juge pénal que dans des hypothèses dans lesquelles le directeur de l'établissement avait commis des manquements très graves mettant en cause sa capacité à respecter le droit à l'éducation. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Centre national d'enseignement à distance (CNED), ou privés -, qui ne sont pas mentionnés dans le texte, afin de maintenir un régime de déclaration pour ces organismes. Pour éviter qu'un simple certificat médical permette d'inscrire son enfant dans n'importe quel organisme d'enseignement à distance, potentiellement douteux ou opérant depuis l'étranger dans la plus grande opacité, il faut distinguer les organismes sérieux, qui ont souscrit à la charte des valeurs et principes républicains, des autres. Pour ce faire, le présent amendement vise à instaurer un agrément, qui pourra être délivré aux organismes d'enseignement à distance hors contrat ayant souscrit à la charte des valeurs et principes républicains, dont les conditions de délivrance seront liées à la conformité de l'enseignement dispensé au socle commun des connaissances ainsi qu'au contrôle de l'obligation scolaire et de l'assiduité des élèves. Quel est l'avis de la commission

ou l'établissement secondaire, en bonne application du principe de subsidiarité et du respect des rôles des parents et de l'école en matière éducative, par la signature, entre l'établissement scolaire et les parents ou les représentants de l'enfant, d'une charte éducative de confiance. Cette disposition contribuerait à lutter contre les démarches séparatistes de certaines familles, dont les enfants sont inscrits à l'école. En effet, l'article L.

111-2, « l'État garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles ». Cet amendement tend donc à formaliser, dans une charte éducative de confiance, le rôle que le code de l'éducation attribue aux parents.

De fait, les places étant limitées, la mobilité restreinte et les codes scolaires inégalement maîtrisés, cette prétendue liberté ne pouvait, en vérité, être exercée que par quelques-uns.

aujourd'hui, politiquement possible ; soyons honnêtes, beaucoup refuseraient. François Dubet et Marie Duru-Bellat le rappellent d'ailleurs dans un ouvrage récent : « Nous condamnons les inégalités scolaires et la reproduction tout en les creusant par nous-mêmes, dès que nous le pouvons. » En matière de mixité dans le secondaire, attention également à ne pas faire de l'État le seul acteur ; il y a, pour les collèges, les conseils départementaux et, pour les lycées, les régions. Il est utile de le rappeler à l'approche des élections ... Par cet article, nous entendons mieux associer toutes les parties prenantes et impliquer les établissements publics et privés ; oui

car, nous ne pouvons pas le nier, ces contrôles sont trop espacés dans le temps. Nous le savons, en cinq ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Il me paraît également important de préciser que c'est au bout de cinq ans d'existence que ces établissements peuvent passer sous contrat, c'est-à-dire après un seul contrôle.

M. Max Brisson. Cet amendement vise à prévoir que l'autorité compétente en matière d'éducation motive sa décision de ne pas octroyer un contrat d'association à une ou plusieurs classes d'un établissement ou d'une école privée. Quel est l'avis de la commission

la commission a émis un avis défavorable de refus de contractualisation entre l'État et une ou plusieurs classes d'une école privée hors contrat soient motivées et qu'elles puissent être contestées devant le juge administratif. Ces exigences de motivation sont applicables en l'état actuel des textes. En effet, ces décisions sont créatrices de droits et, à ce titre, doivent répondre aux exigences de droit commun applicables aux décisions administratives, sans qu'il soit besoin de le préciser dans la loi.

parole est à M. Daniel Salmon. L'article L. 151-4 du code de l'éducation prévoit la possibilité, pour les collectivités territoriales, de verser une subvention aux établissements scolaires privés sous contrat du second degré. Cette disposition issue de la loi Falloux de 1850 représente une ressource importante pour les établissements privés, puisque la subvention peut atteindre 10 % des dépenses annuelles d'une structure. L'ambition du projet de loi que nous examinons aujourd'hui est de lutter contre le séparatisme. Or l'enseignement privé

Nous le savons, la réussite globale dépend de la cohabitation des classes sociales dans les établissements éducatifs. Dès lors, afin de lutter contre le séparatisme social, il nous semble opportun de permettre de conditionner les aides et subventions versées, par les collectivités, aux établissements privés à des objectifs d'amélioration de la mixité sociale et d'origine. L'enseignement privé sous contrat a un rôle à jouer dans cette mixité. L'argent public issu des contributions de la collectivité, donc des citoyens, doit être utilisé pour réduire les inégalités sociales et scolaires.

remettrait en cause l'autonomie des collectivités territoriales et leur liberté d'attribution des subventions. Il faut également noter que le droit encadre déjà fortement les modalités de participation des collectivités territoriales au financement des établissements privés sous contrat.

La mixité dans les établissements scolaires publics est désormais ancrée dans les valeurs de la République ; elle s'est imposée, petit à petit, depuis les années 1960, et a été rendue obligatoire par la loi du 11 loi Haby. Pourtant, presque cinquante ans plus tard, il existe encore plusieurs dizaines d'écoles privées non mixtes. Depuis 2008, il est inscrit à l'article 1 de notre Constitution que la loi prévoit un égal accès des femmes et des hommes à toutes les responsabilités professionnelles et sociales. Il doit en être ainsi de l'accès à un établissement scolaire. Aussi, puisque, depuis quinze jours, les réunions non mixtes retiennent notre attention, je vous demande, mes chers collègues, de mettre fin à cette discrimination anormale dans nos établissements scolaires, en votant cet amendement.

degré. En outre, le directeur d'établissement doit avoir une expérience minimale de cinq ans en tant que professeur ou surveillant d'un établissement scolaire. Or, sur le terrain, certains se jouent de ces règles en inscrivant officiellement, comme directeur, un prête-nom, qui n'assume, dans les faits, aucune responsabilité. Le contrôle académique peut parfois révéler que cette personne n'est même pas présente sur place ! C'est aussi une pratique utilisée par ceux qui dispensent ces enseignements ; ainsi, un professeur est parfois enregistré pour trois classes et le constat fait par l'inspection est que, en réalité, ce sont des assistants d'éducation qui prennent la relève et dispensent les cours,

de la culture ? Mme Delattre vient de le dire, cet amendement vise à lutter contre le recours à une personne prête-nom, qui remplit les conditions de diplôme, d'expérience, de nationalité et d'honorabilité pour devenir directeur, mais qui n'est pas le directeur effectif de l'établissement.

Le contrôle de l'effectivité de la délivrance des enseignements est donc déjà consacré par la loi. Pour ce qui concerne la présence effective du directeur, le ministère est déjà très vigilant. En effet, c'est sur ce contrôle que repose la responsabilité de la gestion de l'établissement au quotidien. doit, en particulier, être en mesure d'intervenir rapidement en cas de problème ; cette exigence d'une présence effective du directeur me semble découler implicitement des dispositions législatives issues de la loi Gatel. Nous n'entendons pas pour autant attendre la réalisation des contrôles pour constater l'existence d'un directeur de fait ; c'est ainsi que mes services se sont déjà opposés à la désignation de certains directeurs qui ne présentaient pas la disponibilité suffisante pour assumer la responsabilité de la direction d'un établissement et qui apparaissaient comme de simples prête-noms. Par conséquent, puisque

Pour enseigner, comme contractuel, dans l'enseignement privé sous contrat, il convient d'avoir un diplôme de niveau bac+3 ou de justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée ; en pratique, dans le supérieur, le niveau de diplôme ou de concours est bien plus élevé.

Quel est l'avis de la commission pour les établissements privés hors contrat. En outre, cet amendement pourrait avoir un effet contre-productif, puisqu'il pourrait être perçu comme garantissant aux établissements privés hors contrat un enseignement

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette disposition vient modifier l'article L. 442-1 du code de l'éducation pour le compléter par un alinéa ainsi rédigé : « L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l'amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements. » Si nous ne pouvons que soutenir cette volonté d'encourager la mixité sociale dans les écoles, nous ne saurions tolérer qu'il stigmatise certains enfants dans certains territoires, du fait de leur origine sociale et de leur confession religieuse. Si le Gouvernement entend réellement veiller à la mixité, qu'il s'y attelle autant dans le XVIII arrondissement de Paris que dans le XVI arrondissement ou ailleurs, ou ailleurs, et autant dans le public que dans le privé. Le Gouvernement ne peut pas faire le choix de la mixité à laquelle il souhaite s'adonner, car une fois de plus, de la même manière qu'il n'y a pas un bon séparatisme et un mauvais séparatisme, il n'y a pas non plus une non-mixité tolérable et une non-mixité inacceptable dans les établissements scolaires.

Autant qu'une condition de la République, le dédoublement des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire, le dispositif « Devoirs faits », les stages de réussite et l'augmentation des bourses de collège sont autant de mesures prises depuis la rentrée 2017 pour l'équité sociale et pour combattre les inégalités à la racine. Nous les défendons, de même que les budgets successifs qui viennent soutenir la priorité accordée à l'enseignement primaire, et ce depuis plusieurs années. Cette disposition tend à renforcer les politiques de brassage des élèves en fonction de leur profil social et nous y sommes favorables. Il est nécessaire d'approfondir et d'amplifier les politiques favorables à un égal service en matière d'éducation. Les établissements publics et privés étant concernés, il est nécessaire qu'ils soient impliqués dans ces actions. il est nécessaire qu'ils soient impliqués dans ces actions. Nous soutenons, monsieur le ministre, cette grande politique publique de mentorat-tutorat que le Gouvernement développe avec un budget tout à fait inédit de 30 millions d'euros, saluée par les associations du secteur. Notre groupe pense qu'il s'agit là d'une nouvelle forme d'éducation populaire, pertinente et efficace. Cette politique s'inscrit en effet dans l'ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui oeuvrent à la transformation sociale et politique en favorisant l'émancipation des plus jeunes. des plus jeunes. Pour ne pas demander aux autres ce que nous ne ferions pas nous-mêmes, il nous faut accroître encore et encore l'accueil des collégiens, lycéens et étudiants dans les institutions pour des stages d'orientation professionnelle et citoyens. Les réseaux doivent également être socialement de la culture ? Cet amendement corrige une erreur de référence d'article pour renforcer le rôle des établissements privés en matière de promotion de la mixité sociale. C'est l'article L. du code de l'éducation qui prévoit ce rôle de mixité sociale du service public de l'éducation nationale et non l'article L. 442-1 du code de l'éducation. En revanche, l'amendement inclut les écoles privées sous contrat simple,

Je profite de la discussion de ces amendements pour obtenir une précision de la part de M. le ministre. Dans le cadre de ses travaux, notamment à l'occasion de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance, la commission de la culture s'est montrée particulièrement vigilante à toute mesure coercitive qui serait de nature à porter atteinte à la liberté d'organisation des établissements privés, laquelle procède de la liberté d'enseignement. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer que le but de l'article 24, ainsi que des articles 24 et 24 est de promouvoir des concertations ou des mesures incitatives ?

a été dit durant notre débat, il est très important d'avoir un objectif de mixité sociale dans le cadre de l'harmonie générale des formules de scolarisation de notre pays. La mixité sociale reste un objectif majeur.

Si l'idée de favoriser une concertation de tous les acteurs de l'éducation autour d'objectifs de mixité sociale est louable, l'article 24 du projet de loi était mal positionné dans le code de l'éducation. C'est pourquoi cet amendement tend à modifier la référence au code de l'éducation, afin que la volonté d'amélioration de la mixité sociale soit un des objectifs communs à l'ensemble des établissements publics ou privés

monsieur le rapporteur l'article 24 Je profite de cet amendement pour alerter sur un obstacle connexe à l'augmentation de la mixité sociale dans les établissements privés sous contrat : le coût du périscolaire et notamment de la restauration scolaire. Tout travail portant sur la mixité sociale au sein des écoles privées sous contrat doit inclure

M. Max Brisson. L'article L. 533-1 du code de l'éducation permet aux collectivités territoriales de faire bénéficier de mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'organisation de l'établissement qu'il fréquente. Cet amendement précise que l'amélioration de la mixité sociale est un des objectifs de ces mesures. Il s'agit de mettre en conformité l'article L. 533-1 du code de l'éducation avec la nouvelle de l'article 24 qui précise désormais que la lutte contre les inégalités sociales et territoriales concerne l'ensemble des établissements qui participent au service public de l'éducation et s'effectue en concertation avec les collectivités territoriales. Cette dimension sociale est déjà inscrite à l'article L. 533-1 du code de l'éducation sous la forme d'une possibilité. Il s'agit donc de mettre en conformité les objectifs de cet article avec ceux que nous venons d'établir par la réécriture de l'article L. 111-1. Quel est l'avis de la commission

prévoit déjà la possibilité pour les collectivités locales, les intercommunalités et les caisses des écoles de mettre en place des mesures à caractère social pour tout enfant, sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente.

par un effet contre-productif, de limiter les possibilités d'action des collectivités locales à ce seul critère, alors qu'elles sont actuellement plus larges, totalement ouvertes. Comme l'a précisé le Conseil d'État en 1996, la notion de « mesures à caractère social » de cet article ne se limite pas à celles qui bénéficieraient exclusivement ou principalement à des familles se trouvant dans une situation économique ou sociale difficile. Des distinctions peuvent être faites sur le plan financier par l'attribution des aides aux élèves selon leurs ressources et leurs mérites. Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement

force est de reconnaître que l'école reproduit, et parfois accentue, les inégalités de naissance. Nous avons tous la responsabilité de lutter contre ce déterminisme social. Aussi, cet amendement présenté par notre collègue Rachid Temal propose que la mixité sociale soit un des indicateurs pris en compte pour la définition de toute nouvelle carte scolaire. Pour ce faire, le revenu médian des foyers fiscaux pourrait permettre d'y parvenir. À toutes fins utiles, je dois préciser que cet amendement a été adopté au Sénat en 2019, lors des débats sur la loi pour une école de la confiance. Il me semble

est la proximité géographique. Faire une carte qui tiendrait principalement compte de la mixité sociale conduirait à des aberrations sur les territoires, notamment en termes de déplacement pour les enfants. Par conséquent, l'avis de la commission est défavorable

je suis d'accord. Un rapport de 2012 de Mme Françoise Cartron, ancienne sénatrice de la Gironde, avait déjà établi ces constats et avançait un certain nombre de propositions sur les problématiques de carte scolaire et de ségrégation.

j'approuve une nouvelle fois la proposition que vous faites, à savoir que toute modification de la carte scolaire, à compter de l'entrée en vigueur du texte, doit intégrer un critère de mixité sociale. Il pourrait, d'ailleurs, s'agir d'une politique à trois niveaux. Tout d'abord, permettre une meilleure sectorisation lorsque cela est possible compenser financièrement le défaut de mixité sociale sur la base d'un indice d'entropie partagé par toutes les parties prenantes ; enfin, dépasser « un confinement social territorial » par des politiques de mise en réseau. Le volontarisme à l'oeuvre en faveur du mentorat doit y participer.

en contradiction avec l'article L. 141-6 du code de l'éducation : « Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique.

Si l'article L. 141-6 du code de l'éducation est suffisamment clair, celui-ci est d'ores et déjà renforcé par le règlement intérieur des universités qui interdit les manifestations religieuses. Laissons aux universités l'autonomie dans leur organisation. Cet article est restrictif et inutile, c'est pourquoi nous proposons sa suppression.

philosophiques, politiques et religieuses. Cela fait partie de leur cursus général et de la façon de de se situer dans la société. Permettez-moi d'évoquer à ce titre un souvenir : quand j'étais étudiant à Nanterre, c'est sur le campus, à l'entrée de la cantine, que j'ai acheté ma première traduction oecuménique de la Bible. J'ai encore ce ce volume et je trouvais tout à fait normal que, devant la cantine, des étudiants m'offrent ce choix. Je pense donc très sincèrement qu'il nous faut être extrêmement attentifs

en essayant de concentrer cette activité sur les aumôneries. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je pense que ce n'est pas une bonne solution. La parole est

code de l'éducation selon lequel « l'État prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse », que ce soit dans les établissements du second degré public ou dans les établissements publics d'enseignement supérieur, sans distinction. distinction. Or ce dispositif est de nature à remettre en cause la légitimité des aumôneries pourtant prévues par l'article 1 de la loi du 9 décembre 1905 qui garantit la liberté de conscience et la liberté de culte. En conséquence, le code de l'éducation prévoit la création des aumôneries dans les collèges et lycées publics comme déclinaison du principe formulé à l'article L. 141-2. On notera d'ailleurs que nombre de ces collèges et lycées incluant, par ailleurs, souvent des classes préparatoires de l'enseignement supérieur disposent d'une chapelle, lieu de culte par excellence, souvent classée ou inscrite à l'inventaire des monuments historiques. de même s'agissant des universités, où elles sont souvent plus anciennes. Par ailleurs, d'un point de vue terminologique, la rédaction est très imprécise, puisqu'elle crée la notion d'« activité cultuelle ». Que recouvre cette notion par rapport à l'« exercice public d'un culte

673. Cet amendement tend à supprimer l'article 24 visant à interdire les activités cultuelles dans les lieux d'enseignement. Cet article introduit en commission est en effet insuffisamment précis et source d'ambiguïté, comme le montre le grand nombre d'amendements de suppression ou de précision déposés. Ces imprécisions portent autant sur la nature des activités interdites, alors même que, aujourd'hui, la présence d'aumôneries n'est pas proscrite, que sur le périmètre de l'interdiction qui concerne, en l'état du projet de loi, les « lieux d'enseignement il n'apparaît pas utile de légiférer sur ce point, dès lors que les responsables des établissements publics d'enseignement supérieur disposent déjà des prérogatives leur permettant de réglementer l'exercice et la pratique d'activités cultuelles dans leur établissement et de concilier ainsi la liberté d'information et d'expression des étudiants avec le respect de l'ordre public et du bon fonctionnement du service public. Premièrement, comme cela a été dit par plusieurs d'entre vous, y compris par le sénateur Ouzoulias, adopter

Ensuite, s'agissant des règlements intérieurs des universités, il me semble qu'ils ont une meilleure assise s'ils s'appuient sur le droit. Notre rôle, aujourd'hui, étant de faire le droit, il me semble que si nous inscrivons ce principe dans la loi, les universités auront davantage de force pour écrire leur règlement intérieur et pour aller dans le sens de la loi. Cela me semble être la moindre des choses. S'agissant des aumôneries- je réponds à la fois à Pierre Cuypers et à Pierre Ouzoulias

d'accord. Nous devons refuser la pratique des prières dans les couloirs des universités. Le prosélytisme est une chose. L'exercice du culte dans un lieu inapproprié ne me semble pas acceptable dans notre République.

Nous disposons d'éléments factuels de pratiques du culte dans des endroits inappropriés. Il me semble que ce texte vise à faire reculer le séparatisme partout où c'est possible, en tout cas à envisager les voies et moyens de le faire. En l'occurrence, nous nous donnons les moyens. Je ne sais pas si cela sera suffisant, sans doute pas totalement. Mais si nous n'acceptons pas de faire un pas en ce sens, nous manquons à notre devoir s'agissant de ce texte. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur ces quatre amendements n 322, 560, 579

... Après deux ans de grève, le pape Grégoire IX, lui-même ancien étudiant à Paris, a édicté la bulle pontificale du 13 avril 1231, qui garantit

La rédaction proposée reste source d'ambiguïtés, notamment du fait de l'emploi des mots « à titre principal ». La suppression de cet article est d'autant plus nécessaire qu'il ne paraît pas utile. En effet, le droit existant permet déjà aux responsables d'établissement public d'enseignement supérieur

Il s'agit bien, ici, de préserver l'ordre public interne des universités. Notre amendement vise donc à substituer aux termes flous d'« activités cultuelles » ceux d'« exercice du culte », qui figurent dans notre législation et qui nous semblent beaucoup plus explicites. Du reste, cette

l'une de théologie catholique et l'autre de théologie protestante. Il existe également un centre autonome d'enseignement de pédagogie religieuse à l'université de Lorraine. En interdisant les activités cultuelles dans les lieux d'enseignement supérieur, cet article faisait peser un risque d'interprétation susceptible de mettre en difficulté les dispositions spécifiques et historiques du droit local. La parole

qui permet l'exercice des cultes. Elle résulte d'un contexte historique, dans lequel la religion catholique était installée

lequel l'exercice des cultes est interdit dans les universités en dehors des aumôneries. Les aumôneries existent, elles sont le produit de l'histoire,

pourquoi je préfère mille fois que nous en restions au droit actuel, ce qui, du reste, ne nous obligerait pas à adopter une disposition spécifique pour nos amis d'Alsace-Moselle.

Une fois encore, il s'agit d'une atteinte à la liberté associative. Elle part d'une suspicion détestable jetée sur le monde associatif, que celui-ci fait vivre notre République, au quotidien, à travers ses milliers de bénévoles. Cet article alourdira considérablement les procédures pour les très nombreuses petites associations étudiantes qui bénéficient non pas forcément de subventions, mais d'une simple mise à disposition de salle. Désormais, une association étudiante de danse ou de chorale devra signer un contrat d'engagement républicain pour bénéficier d'un local au sein de sa propre université. Là où tout était simple et où tout fonctionnait bien, vous instaurez la défiance. Vous introduisez une lourdeur administrative, alors que tout au long de l'année vous êtes d'habitude si nombreux à dénoncer Croyez-vous réellement que la radicalisation opère dans les clubs d'échecs ou les tournois de volley à l'université ? Pour toutes ces raisons, je vous invite à faire preuve de modération, mes chers collègues, et à supprimer cet article.

sur la mise à disposition de locaux qui pourrait être considérée comme une subvention en nature et donc conditionnée à cette souscription. Les auditions des représentants du monde universitaire

appliquée depuis vingt ans entre les collectivités territoriales et le mouvement associatif, nous souhaiterions en étendre l'application aux établissements publics d'enseignement supérieur. Depuis 2001, la charte des engagements réciproques a été signée entre l'État, les représentants des associations de collectivités et ceux du mouvement associatif. Rénovée en 2014, elle a déjà été étendue de façon sectorielle au ministère de la justice en 2015, les signataires étant la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et les associations oeuvrant

démontre le besoin d'éviter toutes les dérives incompatibles avec les principes fondamentaux du service public, de citoyenneté et d'égalité devant la loi. Nul ne peut se prévaloir de la liberté d'expression ou prétexter d'un quelconque respect des identités ou des races pour porter atteinte à ces principes.

d'exercer des pressions sur les membres de la communauté universitaire ou de perturber, par du prosélytisme ou de la propagande, l'enseignement, la recherche ou les conférences et débats autorisés par le président de l'établissement. Nous avons du mal à comprendre l'intérêt de ce dispositif qui complète l'article L. 811-1 du code de l'éducation, pourtant déjà très explicite. En effet, le code de l'éducation prévoit actuellement que les usagers du service public d'enseignement supérieur disposent de la liberté d'information et d'expression sur les problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, et qu'ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.

Ne nous y trompons pas, il s'agit là du retour de l'article 38 de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, censuré par le Conseil constitutionnel il y a quelques mois ! Que nous dit cet article, sinon que la liberté d'information et d'expression des usagers du service public de l'enseignement supérieur ne saurait leur permettre d'exercer des pressions sur les autres membres de la communauté universitaire, d'avoir un comportement de nature à perturber par des actions de prosélytisme ou de propagande les activités d'enseignement et de recherche, la tenue de conférences ou de débats autorisés par le président d'université ou le directeur de l'établissement, ou de troubler le bon fonctionnement du service public

Cet amendement s'inscrit dans la lignée des mesures antisyndicales qui criminalisent le mouvement social étudiant. Dans la droite ligne des lois portées par le Gouvernement depuis quelques mois, il acte une fuite en avant répressive. La démocratie étudiante est un espace précieux de citoyenneté et d'émergence de liberté. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. La

les dispositions de l'article L. 811-1 du code de l'éducation permettent déjà aux responsables des établissements publics d'enseignement supérieur de concilier la liberté d'information et d'expression des étudiants avec le respect de l'ordre public et du bon fonctionnement du service public. La portée des dispositions a, par ailleurs, déjà été précisée par le Conseil d'État, notamment dans une décision du 26 juillet 1996 que se borne à reprendre l'article 24 . Le risque est grand que les acteurs de l'enseignement supérieur ne voient dans ces nouvelles dispositions un infléchissement du droit en vigueur, alors qu'elles se bornent à le confirmer.

La liberté d'information et d'expression des usagers du service public de l'enseignement supérieur, notamment des étudiants, fait effectivement partie des libertés fondamentales des universités : personne ne le conteste. La décision du Conseil d'État, en 1996, qui a servi de base à la rédaction de cet article, autorisait, en l'espèce, les jeunes filles à aller en cours en portant un voile.

Certes, l'université est un lieu d'enseignement, de recherche et de débat, mais il faut permettre qu'elle le reste. Je ne comprends donc pas la réticence à inscrire dans la loi des interdictions. Monsieur le ministre, vous venez de dire que la mesure est d'ordre réglementaire, et qu'un règlement intérieur peut suffire à poser ce genre d'interdits.

qui perturbe et qui nuit aux activités de recherche et d'enseignement sera interdite, puisqu'elle sera caractérisée et identifiée dans la loi. Quant aux « troubles à l'ordre public », ils feront l'objet de l'amendement suivant, que je vous présenterai

le débat que nous tenons est très symptomatique des impasses auxquelles conduit votre volonté absolue. Vous dites qu'il faut lutter contre le djihadisme violent et ses ravages, et vous avez raison. Cependant, vous pensez que, pour atteindre ce but, nous devons entrer dans des quantités de considérations, de règles en tout genre, qui n'auront pas d'effet sur l'objet visé.

M. le rapporteur pour avis : empêcher quelqu'un de parler dans une université, c'est scandaleux, c'est horrible, et on ne doit pas l'accepter. Cependant, qui doit agir ? Sur ce point, je rends hommage à Pierre Ouzoulias, parce que, depuis le début de ce débat, il nous dit que la question centrale ce sont les franchises universitaires.

modèle des universités hongroises où la liberté d'expression et le débat sont interdits ? Vous savez bien que c'est dans les universités que sont nées les grandes théories et les grandes réflexions,

Encore une fois, à force de caricaturer, on oublie l'essentiel : nous sommes tous contre l'islam radical dans sa manifestation totalitaire- c'est une évidence.

Revenons un peu à ce qui nous réunit ce soir, puisque nous sommes en train de faire la loi. Aujourd'hui, il faut concilier à la fois la liberté d'information et d'expression des étudiants et le respect de l'ordre public.

Alors, ne montons pas en épingle les manifestations de quelques étudiants, qui ont effectivement empêché certaines célébrités de venir s'exprimer dans un amphithéâtre ! Ce n'est pas cela, l'université. Si nous nous concentrons sur notre travail de législateur, l'article 24 n'est pas nécessaire. S'il était adopté, il imposerait une conception de l'université

est absurde dans le sens où ces professionnels travaillent les uns et les autres dans les mêmes unités mixtes de recherche. Il est anormal qu'ils ne disposent pas des mêmes garanties. C'est pourquoi je vous propose d'unifier et d'homogénéiser ces régimes de protection en étendant aux chercheurs du CNRS, par exemple, les droits des enseignants-chercheurs de l'université.

à ce sujet. Pourriez-vous nous apporter des éléments qui seraient de nature à les rassurer, monsieur le ministre, et notamment confirmer que l'article L. 411-3 du code de la recherche offre les mêmes garanties aux chercheurs que l'article L. 952-2 du code de l'éducation ? Quel est l'avis du Gouvernement ?

: « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité.

M. Max Brisson. Depuis plusieurs années, on assiste au développement de revendications communautaristes, le plus souvent à caractère religieux, au sein de certaines listes électorales candidates aux élections des représentants des étudiants. Cette montée du communautarisme religieux relève d'un prosélytisme qui doit être rejeté sans ambiguïté, car il va à l'encontre de la tradition laïque de l'université française. Aussi le présent amendement vise-t-il à empêcher la présence de listes communautaristes lors des élections organisées au sein des établissements universitaires. de la culture ? Je partage l'avis et la démarche de Max Brisson pour lutter contre la montée du communautarisme. On constate dans certaines universités la présence

l'Union des étudiants juifs de France, l'Union générale des étudiants de Tunisie, l'Union des étudiants créoles dans telle UFR de telle université, l'union de telle ou telle contrée, autant de listes qui pourraient remettre en cause le caractère un et indivisible de la République en raison d'un régionalisme

vous n'avez fait aucun pas, me semble-t-il, vers ceux qui luttent contre le communautarisme. Je vous le disais en m'emportant- paraît-il -la semaine dernière, je vous le dis cette fois très calmement : vous trouvez toujours une bonne raison

qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public ». Le port de signes Le port de signes ou de tenues ostentatoires manifestant une appartenance religieuse peut constituer un moyen de pression sur le corps enseignant sur la liberté de conscience des autres étudiants, en contradiction avec l'article L. 141-6 du code de l'éducation Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à interdire à l'université le port de signes qui manifestent de façon prosélyte l'adhésion à une opinion religieuse, politique ou philosophique.

enseigner, organiser des conférences, faire vivre l'université comme lieu de recherche et de débat à l'abri des pressions de tout ordre : nous avons évoqué ces enjeux tout à l'heure. Nous avons précisément adopté un article visant à encadrer cette liberté d'expression

C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Monsieur Bascher, je vous félicite : vous avez anticipé leur demande, car votre amendement tend à supprimer toute forme d'enseignement religieux en Alsace-Moselle ; c'est brillant

cette interdiction ? C'est M. Erdogan, pour arriver, non pas à l'islamo-gauchisme, mais peut-être à un islamo-fascisme propre à la Turquie. la Turquie. On peut dire ce que l'on veut ; voilà la réalité de l'histoire ; voilà la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Monsieur le ministre, vous vous en souvenez peut-être et Max Brisson le sait parfaitement